Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les mesdames, messieurs les sénateurs, avant toute chose, je souhaiterais saluer celles et ceux- ils sont nombreux dans cet hémicycle -qui, depuis le début de l'examen de ce texte, et même depuis de très longs mois, ont été au rendez-vous afin d'adopter les mesures que les circonstances exigeaient pour protéger la santé de nos concitoyens, dans des conditions souvent difficiles. Par-delà les désaccords, par-delà les divergences, je sais combien le Sénat est engagé dans la lutte contre l'épidémie. La commission mixte paritaire qui s'est tenue jeudi dernier s'est toutefois soldée par un échec, duquel personne ne sort gagnant. Il nous appartient désormais de poursuivre et d'achever l'examen du texte, en gardant intacte notre exigence de protéger les Français face à un virus qui circule à très grande vitesse et qui a déjà entraîné tant de morts et de sacrifices. Le débat est indispensable, et rares sont les pays du monde qui, face à cette pandémie, ont accordé autant de temps et d'importance au débat démocratique. La première lecture a d'ailleurs prouvé que nous pouvions ensemble enrichir ce texte, l'adapter, le modifier et le faire évoluer, pour qu'il soit à la fois équilibré et efficace. Il a été question de « raz de marée ». L'expression n'a rien de galvaudé, puisque nous recensions, hier encore, plus de 300 000 nouveaux cas, 24 000 hospitalisations et 3 500 patients en soins critiques. Cette situation sans précédent demande du sang-froid et exige que nous prenions nos responsabilités en vue de poursuivre la gestion d'une épidémie toujours virulente, qui dure depuis bientôt deux ans. Pour y faire face, le projet de loi renforce plusieurs mesures existantes qui nous ont d'ores et déjà permis de contenir l'épidémie et d'éviter les choix plus radicaux auxquels plusieurs pays européens ont été contraints en raison de décisions différentes dans la gestion de la crise. Je ne reviendrai pas sur les lignes de force d'un texte qui vous a déjà beaucoup mobilisés ; je rappellerai simplement que celui-ci s'appuie sur ce que nous savons du virus et sur ce dont nous disposons pour le combattre efficacement. Aujourd'hui, malgré la présence d'un variant extrêmement contagieux, si nous pouvons envisager de vivre le plus normalement possible, sans empêcher ou fermer massivement les activités du quotidien, c'est parce que nous avons un vaccin. Et celui-ci permet d'éviter, dans l'immense majorité des cas, de développer des formes graves de la maladie. Il nous faut poursuivre nos efforts de persuasion et aller vers celles et ceux qui, tantôt par indifférence, tantôt par éloignement, tantôt par une défiance qui dépasse parfois l'entendement, n'ont pas encore franchi les portes d'un centre de vaccination. J'en viens au texte que nous remettons sur le métier. Malgré l'échec de la commission mixte paritaire, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale et qui vous a été transmis reprend plusieurs apports importants du Sénat. Je pense tout d'abord aux améliorations concernant la possibilité d'application du passe sanitaire aux réunions politiques, aux conditions de recours cumulatif au passe vaccinal et à la présentation du résultat d'un test de dépistage. Je pense aussi à la reprise des travaux du Sénat visant à préciser et à simplifier les modalités d'application du passe aux mineurs, permettant d'aboutir à un équilibre sur ce sujet, qui tenait à coeur à de nombreux parlementaires. Je me réjouis de nouveau de l'adoption de dispositions en première lecture, permettant d'appliquer aux mineurs de 5 ans à 11 ans les règles applicables à leurs aînés en matière d'autorisation parentale, afin de faciliter le déroulement des opérations de dépistage et de vaccination. pourrais citer aussi la sécurisation du pouvoir d'adaptation des nouvelles règles par les préfets, notamment outre-mer, lorsque les circonstances locales l'exigent. J'aimerais également mentionner les précisions apportées quant aux modalités de contrôle du passe, qui avaient été adoptées en commission sur l'initiative de votre rapporteur, avant qu'elles ne soient supprimées en séance. L'Assemblée nationale a toutefois repris ces améliorations, afin de lever les inquiétudes qu'avait pu susciter le dispositif relatif à l'identité des personnes lors de la présentation du passe. La suppression de toute disposition à ce sujet et celle du dispositif de sanctions administratives des entreprises ne respectant pas leurs obligations de prévention, malgré les ajustements adoptés en nouvelle lecture sur le niveau des sanctions pour assurer leur proportionnalité,

Malgré les discussions menées sur ces deux points jusqu'à la commission mixte paritaire, je constate en l'état que les désaccords persistent. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le voyez, ce texte a été discuté largement et enrichi par les travaux de chaque assemblée. Le projet de loi qui vous a été transmis est un texte équilibré, adapté à la gravité des circonstances autant qu'à l'exigence démocratique qui ne nous a jamais quittés, ainsi qu'à la protection des libertés individuelles dans un contexte de menace sanitaire sans précédent. La situation requiert donc que nous dépassions nos divergences pour nous hisser collectivement à la hauteur de ce défi sanitaire. Je ne doute pas que, au-delà des désaccords de fond, nous poursuivrons avec cet esprit de responsabilité. La parole

Le 27 décembre dernier, le conseil des ministres adoptait un texte qu'il avait soumis la semaine précédente au Conseil d'État. Depuis Depuis cette date, que d'évolutions ! Le 27 décembre, que savions-nous du variant omicron ? Peu de choses en vérité.

sur les admissions en services de soins critiques et sur les hospitalisations. Certes, la courbe continue à progresser dans le mauvais sens, mais force est de constater que la flambée sans précédent

de l'épidémie causée par ce coronavirus. Il existe une possibilité, qui n'est pas encore une certitude, pour que, après avoir évincé

qui viennent. Pour apprécier la portée du vote que je vais vous proposer de confirmer, je souhaite que le Sénat mobilise toutes les ressources de ses moyens d'évaluation des politiques publiques, de ses moyens de contrôle

a bien sûr exprimé des interrogations et des doutes. Ce qui lui importe, c'est que, en contrepartie de son acceptation du passe vaccinal, le contrôle parlementaire ait lieu.

mixte paritaire ont été ... ce qu'ils ont été.

un constat d'échec que rien ne laissait augurer. En effet, nous en étions parvenus à l'examen des rédactions traduisant l'accord politique qui avait été conclu

de la représentation nationale sur le principe du passe sanitaire. Cette disposition d'esprit, qui est celle de la commission des lois, connaît seulement deux limites, mais qui sont essentielles.

force est de constater que sur ce texte important, qui vise l'objectif de consolider l'arsenal de la lutte contre l'épidémie, et ainsi de protéger la santé des Français, nos positions n'étaient pas si éloignées. porte la marque des efforts déployés par Chantal Deseyne et Philippe Bas pour tenter de parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Sur les articles pour lesquels notre commission a reçu une délégation au fond- différents articles additionnels relatifs à l'organisation des soins ou au droit du travail, ainsi que l'article 3 prévoyant une saisine systématique du juge dans le cadre du renouvellement des mesures d'isolement et de contention en services de soins psychiatriques sans consentement je regrette que, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'ait, pour l'essentiel, pas retenu les différentes améliorations proposées par notre commission concernant l'encadrement de la prise en charge des téléconsultations, l'aménagement des reports des visites médicales en santé au travail ou encore visant à une rédaction plus protectrice de l'article 3. Cependant, la commission des affaires sociales a considéré que, dans le contexte d'urgence dans lequel nous nous trouvions, il était de notre responsabilité de favoriser une entrée en application rapide du passe vaccinal et que cette nouvelle lecture ne devait pas rouvrir l'ensemble des discussions que nous avions pu avoir cette semaine. Notre attention s'est ainsi focalisée sur l'un des principaux points de divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui est, en matière de droit du travail, le régime de sanction administrative applicable aux employeurs qui ne respecteraient pas les principes de prévention des risques d'exposition de leurs salariés à la covid-19. Notre commission avait supprimé cette disposition en première lecture lors de l'examen du projet de loi en séance publique, le Sénat a aussi très largement repoussé la proposition du Gouvernement de rétablir l'article 1 A. L'Assemblée nationale a rétabli cet article, avec pour seule modification la réduction du montant maximum de l'amende due par les entreprises en cas de manquement constaté à la protection de leurs salariés face à la covid-19, de 1 000 à 500 euros par travailleur. Ce n'est pas satisfaisant. Cette concession symbolique de l'Assemblée nationale, si elle atténue quelque peu la nocivité du dispositif, est loin de répondre aux réserves de principe du Sénat. Nous l'avions dit, ce nouveau régime de sanctions n'est ni souhaitable ni utile. Cette logique coercitive ne correspond pas à la mobilisation des entreprises depuis le début de la crise sanitaire pour assurer la santé et la sécurité de leurs salariés dans le contexte épidémique. Force est de constater, comme l'a montré l'intervention de la ministre du travail mercredi soir, que cet article se borne à servir la communication du Gouvernement sur le recours au télétravail, sans renforcer la protection de la santé des travailleurs. Comment expliquer, sinon, qu'après avoir communiqué sur une sanction de 1 000 euros pour les entreprises qui ne se conformeraient pas aux recommandations de trois jours de télétravail, la ministre nous indique au banc du Gouvernement qu'il n'est nullement question de télétravail dans cet article La commission a donc réaffirmé son opposition au dispositif de sanctions et a, une nouvelle fois, supprimé l'article 1 A. Vous l'aurez compris, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a suivi une position claire et responsable oui au passe vaccinal, selon des contours améliorés grâce au travail de notre commission des lois ; non à une mesure inutile d'immixtion de l'inspection du travail dans la gestion du télétravail par les entreprises. La parole

Dossus. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comment en sommes-nous arrivés là ? Comment sommes-nous passés d'un texte d'urgence, qui devait quasiment être voté entre Noël et le jour de l'an, à un combat politicien entre le Gouvernement et la droite sénatoriale ? Pour cela, il a fallu que chacun y mette du sien ! De l'arrogance gouvernementale, il y en a eu, beaucoup, allant même jusqu'à l'insulte et la vulgarité, ce gouvernement mettant dans le même sac les désinformateurs et les désinformés. Le même gouvernement qui justifiait, il y a quelques semaines, l'urgence d'un nouveau texte par l'objectif de sauver des vies a décidé cette fois de prolonger les débats, trouvant un prétexte grotesque pour faire échouer la commission mixte paritaire ! Tout au long des débats, les oppositions étaient- je cite le Gouvernement -« irresponsables » de déposer des amendements, de questionner ses choix ou de s'opposer au principe même du passe vaccinal. Pendant ce temps, deux ans après le début de cette pandémie, l'hôpital est toujours sous pression extrême et ne tient que par le dévouement de son personnel au bord de l'épuisement. Pendant ce temps, l'éducation nationale subit toujours le mépris et le dilettantisme de son ministre. Pendant ce temps, la circulation massive du virus ne faiblit pas. Pendant ce temps, les Françaises et les Français sont fatigués par le niveau de leurs représentants. Néanmoins, pour se vautrer dans la politique politicienne, le Gouvernement n'était pas seul. Il a trouvé ici des partenaires de choix. Le tweet du président Retailleau va pouvoir rejoindre les annales de l'histoire parlementaire. Pour la première fois, une commission mixte paritaire, partie pour trouver un difficile accord, a échoué à cause d'une expression malheureuse sur Twitter. La droite sénatoriale s'est montrée plus intéressée par sa campagne présidentielle que par la crise sanitaire La gestion de la pandémie ne devrait pas se résumer à une bataille puérile entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ou entre La République En Marche et Les Républicains. Cet épisode peu glorieux a mis à nu l'objectif politicien qui sous-tend ce texte. ce texte. Il ne fera qu'alimenter l'antiparlementarisme dans notre pays. C'est désolant ! La situation nécessite davantage de maîtrise de soi, de recul et de hauteur de vue, mais telle n'est décidément pas la tonalité politique du moment. Nous appelons à l'humilité face à la difficulté de la tâche qui est la nôtre. Si nous avons contesté certains des choix opérés, nous avons toujours proposé d'autres voies pour faire face à la situation. Oui, la vaccination massive de la population est indispensable. Saluons d'ailleurs l'adhésion d'une très grande majorité de Françaises et de Français au vaccin et aux rappels. Oui, la vaccination protège. Oui, il faut continuer de convaincre et d'aller vers les publics non vaccinés, y compris les plus réfractaires, pour les amener à se vacciner.

Le tout-numérique comme mode d'organisation, par exemple, remet en cause l'égalité de l'accès aux soins. Un autre phénomène se maintient dans le temps : celui de la forte corrélation entre le niveau de pauvreté des habitants d'une commune et le taux de non-vaccination.

une politique de prévention sanitaire et de dialogue avec les élus locaux et la société civile est plus efficace que la multiplication de mesures globales coercitives. Aussi, notre groupe propose que l'État assume son rôle et contribue sincèrement à la protection des personnes, en mettant à disposition des publics exposés des masques FFP2, plus protecteurs contre la propagation du covid, et en fixant leur prix par décret. J'ajouterai un dernier mot sur le variant omicron. Celui-ci ne sort pas de nulle part. Il n'est pas une catastrophe naturelle ! Il est la conséquence d'une circulation accrue du virus dans des parties du monde où la vaccination n'atteint pas les taux que nous connaissons dans notre pays. Tant que nous ne ferons pas des vaccins un bien public mondial qui puisse être produit massivement à moindre coût sur tous les continents, nous serons susceptibles de connaître des vagues futures de contaminations et d'autres d'échappements immunitaires. La France doit être au rendez-vous et appuyer toutes les démarches qui vont dans le sens d'une levée des brevets. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous nous opposons à la philosophie générale de ce texte, à l'instauration d'une société de contrôle, punitive et infantilisante, à l'instrumentalisation politique de cette crise par le pouvoir exécutif et aux restrictions de nos libertés qui n'ont que peu d'effets sur la propagation de l'épidémie. Notre groupe demande une autre politique de gestion sanitaire pour endiguer l'épidémie : une vaccination qui n'oublie personne, un moratoire sur les fermetures de lits dans les hôpitaux, la généralisation des capteurs d'air, la gratuité des tests et des masques les plus protecteurs, enfin, le combat pour la vaccination mondiale. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comment ne pas avoir cette après-midi une sensation de déjà-vu ? Après des jours et des jours de « vous allez voir ce que vous allez voir ! », évoquant un Sénat gardien des libertés publiques, raisonnant à l'écart de la pression de l'urgence, vous nous expliquez aujourd'hui, monsieur le rapporteur, que la raison, en définitive, c'est justement de voter le texte du Gouvernement et de l'Assemblée a retoqué pour l'essentiel l'apport sénatorial. Pourtant, monsieur le rapporteur, vous nous avez répété à maintes reprises, depuis plusieurs semaines, que ce texte ne répondait pas à une urgence sanitaire qu'il n'aurait aucun impact sur la vague actuelle. Et qui, à part le Gouvernement, pourrait prétendre le contraire ? Ce que vous nous demandez d'adopter, avec le Gouvernement, c'est un texte anachronique. La stratégie de la restriction des libertés publiques n'a pas marché contre la propagation du virus, ni pour le variant delta ni pour le variant omicron. Bien entendu, la simple annonce du passe sanitaire a provoqué une forte progression de la vaccination, ce dont nous nous félicitons. faut-il se vanter d'avoir recours à la coercition parce que notre système de santé, de l'hôpital à l'assurance maladie en passant par la médecine de ville, est exsangue et n'a pas pu mener par la persuasion une campagne de vaccination, comme ce fut le cas dans de très nombreux pays ?

nous voterons contre ce projet de loi, car il n'a pas lieu d'être sur le plan sanitaire. Mais nous voterons aussi contre ce texte, car, comme ceux sur le passe sanitaire et sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, il participe à la transformation de notre société, à sa fracturation, à sa mise sous coupe. Mes chers collègues, nous n'acceptons pas que l'Assemblée nationale, avec l'assentiment d'une majorité de circonstance, s'assoie sur le vote des 303 sénateurs

Je le répète, cette politique masque la casse de l'hôpital public, la fermeture de lits durant l'épidémie, l'incapacité de notre industrie à produire le vaccin, l'assèchement de la recherche le manque de moyens à tous les étages, notamment à celui de l'école, pour réorganiser la société face à cette terrible crise que nous traversons. Jamais nous n'avons obtenu une discussion sérieuse sur la question clef de la levée des brevets ! Pourtant, nous y adjure. La multiplication des doses de rappel dans les pays riches n'est pas la solution à long terme. Il faut vacciner l'humanité tout entière ! Tout à fait ! Enfin, mes chers collègues,

Mercredi soir, nous avons rappelé qu'il est nécessaire de sortir de la gestion sanitaire de la crise décidée par Emmanuel Macron, entouré de son conseil de défense opaque. C'est l'ensemble des acteurs de la société qu'il faut mobiliser, et le Parlement doit reprendre pleinement sa place de décideur. le Parlement, y compris malheureusement le Sénat, accompagne le Gouvernement dans ses choix antidémocratiques à l'efficacité contestable quant à la lutte contre la pandémie. Nous voterons donc contre ce texte dépassé, dont l'objectif est politique et non sanitaire.

Certes nous assistons à une multiplication des doses qui interpelle jusqu'à l'OMS, où l'on s'interroge sur la stratégie française. Mais si cela permet de réduire les formes sévères et d'éviter que le pays ne soit immobilisé en raison de la saturation des services hospitaliers, il faut s'en satisfaire un tant soit peu.

bien ! Même si j'aurais aimé que nous allions plus loin en décidant de sa suppression, le Sénat a encadré son usage avec plus de rigueur. Lors du précédent examen, le groupe RDSE avait présenté des amendements allant dans le sens de l'état de droit. Bon nombre d'entre eux furent d'ailleurs satisfaits.

l'usage du passe dans les transports interrégionaux. Notre commission avait adopté un dispositif introduisant une souplesse attendue, et nous avions poursuivi cet assouplissement en séance. Dans le même esprit, les propositions de notre rapporteur fixaient davantage de limites et encadraient plus strictement ce passe. Nos débats en séance publique avaient participé à réduire encore son champ d'application et à supprimer certains de ses effets particulièrement nuisibles.

des citoyens se sentent mis au ban et des entreprises sont fragilisées. Eh oui ! Il y avait, de mon point de vue, d'autres moyens de protéger sans exclure. Après la mobilisation populaire, même les légères adaptations décidées en toute

J'alerte donc de nouveau les pouvoirs publics, car il y a une lame de fond contestataire, que la ministre de la mer, complètement déconnectée de nos réalités locales, n'a pas anticipée, pas plus que d'autres élus il est vrai. Cela va bien au-delà des appartenances politiques : il s'agit d'un problème bien plus profond. Par manque de courage politique au niveau national, nous sommes passés à une société d'exclusion qui brise définitivement le contrat social de Rousseau, ce qui est profondément choquant de mon point de vue. C'est un changement de paradigme que nombre de décideurs publics n'ont pas perçu sur la durée.

ce passe a tant de conséquences sociales désastreuses, notamment dans un petit territoire comme le mien, qu'il faudra encore l'assouplir sans attendre la clause de revoyure annoncée par l'État comme une espèce de carotte, qui revient à infantiliser nos compatriotes. Ce n'est pas cela, le contrat social ! Aussi, vous l'aurez compris, je voterai contre ce texte, même si le groupe RDSE dans sa majorité se prononcera favorablement. La parole est

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi de vous dire que vous êtes le Gouvernement du retard Vous avez été les derniers à fermer les frontières, les derniers à fournir des masques aux soignants, les derniers à prendre au sérieux l'épidémie. Mais vous êtes aussi les derniers à croire que le masque sert à quelque chose dans la rue, les derniers à restreindre les libertés pour lutter contre un variant très peu virulent, les derniers à estimer que seule la vaccination nous sauvera, les derniers à penser que nous n'atteindrons jamais La « start-up nation » vantée par Emmanuel Macron ressemble plutôt à la « soviétique-nation », et le « nouveau monde » est pire que l'ancien : des rouages rouillés et des « emmerdements » en pagaille. Même les communistes de cette assemblée vous trouvent liberticides, c'est dire L'opposition de droite dans cet hémicycle est pétrifiée, parce que la parole des vrais opposants est diabolisée. Ceux qui sont favorables au passe vaccinal sont des gens responsables, ceux qui s'y opposent sont des irresponsables, des antivax, des sous-citoyens. Nous n'avons même pas le droit de dire ou de penser qu'une autre voie est possible. Regardez pourtant le taux d'incidence est certes élevé, mais il reste sans commune mesure avec le faible taux de létalité. C'est au moment où l'épidémie est la moins grave que vos contraintes sont les plus fortes. Cette disproportion n'a d'égale que votre déconnexion. Ou alors, vous cherchez à entretenir la psychose en vue de cacher le calamiteux bilan de votre quinquennat. Ce gouvernement par la peur est illégitime. Avant 2020, les plans blancs déclenchés en situation de crise dans les hôpitaux avaient lieu chaque année, sans passe vaccinal ou passe sanitaire. Tout cela nous est infligé depuis des années parce que vous avez volontairement réduit l'hôpital à l'os. Avec ce passe, vous ne réglerez ni le problème de l'épidémie, ni les déprogrammations d'opérations en cascade, ni les retards pris dans le diagnostic de nouvelles maladies graves. À l'heure où tout le monde change de braquet, vous vous obstinez. Regardez l'Espagne : les efforts ont été concentrés sur les personnes à risques, et le Gouvernement ouvre le débat sur un grand retour à la normale. A-t-on le droit d'avoir ne serait-ce que ce débat ici même ? Nous avons eu un ministre triple vacciné et contagieux dans cet hémicycle il y a deux jours. Nous n'en ferons pas un bouc émissaire, mais cela doit rappeler toute notre assemblée au bon sens et inviter le Gouvernement à l'humilité. Pour ma part, Gaulois réfractaire non vacciné, non antivax mais prolibertés, je me suis fait tester ce matin. Je suis en bonne santé et je ne fais pas la leçon aux vaccinés qui tombent malades, car je refuse de tomber dans le piège de la surveillance généralisée et de la division des Français. J'observe uniquement que les décisions graves que vous prenez sont dictées par une stratégie et un objectif politique et non sanitaire. Le coût direct de vos restrictions et de vos contraintes aurait pu servir à un investissement massif en personnel et moyens dans l'hôpital. Chers collègues, en tant que citoyens et parlementaires, nous devons garantir le respect des droits, protéger la liberté et la santé de nos compatriotes. À l'école de Montesquieu, je crois que « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. » C'est pourquoi je serai de nouveau présent cette après-midi pour prendre part aux débats et m'opposer, encore et toujours, à ce passe vaccinal.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre groupe a toujours défendu dans ce débat une position claire : l'obligation vaccinale.

Cela dit, nous avons vécu quelques péripéties depuis lundi dernier et nous comprenons qu'un certain nombre de nos concitoyens aient du mal à s'y retrouver.

Aussi ai-je été un peu surpris d'apprendre qu'un accord putatif, dont je n'ai d'ailleurs jamais eu connaissance, aurait été élaboré avant l'événement extérieur dont nous avons parlé. J'en profite pour dire que nous sommes envahis par une société du virtuel, en particulier en politique. Or,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il ne me paraît pas difficile, à ce stade de la procédure législative, de rétablir les bases du débat

de lutte contre la pandémie et de protection de notre population- un outil supplémentaire -et qu'il ne fallait pas tarder à l'instaurer. Il y avait,

par le Conseil d'État avant la présentation du projet de loi et qui s'applique tout à fait couramment et sans mise en cause des libertés, que ce soit pour payer une dépense par chèque ou pour acheter un paquet de cigarettes quand on paraît jeune. En

alors que cette méthode de contrôle et de sanction figure dans le code du travail depuis des décennies et qu'elle est pratiquée avec mesure par l'inspection du travail, sous un contrôle hiérarchique puis juridictionnel qui élimine tout risque

au profit, parfois, de formules de compromis heureuses, comme l'abaissement du plafond des sanctions prononcées par les inspecteurs du travail ou l'instauration du caractère facultatif de l'exercice du contrôle de conformité.

ou peut-être envisager de tromper son auditoire, que de prétendre que ce caractère facultatif prive de toute efficacité le contrôle de conformité. Je veux y insister, mes chers collègues, rien que le travail de police- Dieu sait qu'il est difficile

passes vaccinaux visiblement frauduleux et qu'ils appliqueront, même si c'est de façon volontaire et facultative, cette

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lors de l'examen du texte sur le passe vaccinal en première lecture, nous avons été à la fois amusés et consternés par les péripéties intervenues à l'Assemblée nationale. Notre chambre, quant à elle, a terminé avec sérieux l'examen du projet de loi, à une heure tardive, dans la nuit de mercredi à jeudi. Nos efforts auront pourtant été, vous en conviendrez, mes chers collègues, bien mal récompensés, car, au moment où un accord sur le texte se dessinait enfin en commission mixte paritaire, patatras ! Nous voilà donc réunis en ce samedi après-midi, avec bien moins d'espoir de faire entendre la voix du Sénat. Ce texte est pourtant capital pour les mois à venir. Nous avons tous en tête le nombre record de contaminations quotidiennes dans notre pays et nous gardons les yeux rivés sur le taux d'occupation des lits de réanimation. Cette pandémie dure depuis maintenant près de deux ans. Nos soignants sont exténués, tout comme le reste de nos concitoyens, mais ils sont aussi conscients que la gestion française de la crise sanitaire est parmi les meilleures au monde. Notre pays a beaucoup souffert, mais le Gouvernement et le Parlement ont fait en sorte de préserver, le mieux possible, la santé et la liberté de nos concitoyens. Nous avons aussi protégé au maximum notre tissu économique et l'éducation de nos jeunes. Aujourd'hui, à l'heure de la cinquième vague, très peu de lieux sont fermés en France et nos concitoyens n'ont pas eu à subir de nouveaux confinements, à la différence des citoyens des Pays-Bas ou encore de l'Autriche. Même si la vigilance reste de mise, nous devons cette situation favorable à un miracle : le vaccin. Rien ne permettait de penser que celui-ci serait mis au point aussi rapidement et rien ne garantissait non plus que nous y aurions massivement accès.

Malheureusement, certains, bien qu'éligibles à la vaccination, ont fait un autre choix ; pour des motifs qui leur appartiennent, ils persistent à refuser de se faire vacciner. Ce faisant, ils ne mettent pas seulement en péril leur propre santé, ils menacent également celle des autres. Depuis trop longtemps, nos services de santé sont contraints de déprogrammer des soins. Cela signifie que des Français voient leur traitement reporté afin que des non-vaccinés puissent être soignés. Ce n'est pas acceptable. Pour faire société, nous devons tous être responsables, nous devons répondre des conséquences de nos actes. Le passe sanitaire sera prochainement transformé en passe vaccinal. L'objectif est d'éviter la contamination de ceux de nos concitoyens qui n'ont pas d'anticorps ; à la fois pour préserver leur propre santé, mais aussi pour limiter autant que possible la saturation des services de réanimation. Cette mesure ne fait pas l'unanimité au sein de la société, mais, me semble-t-il, elle divise beaucoup moins qu'on ne le croit. La grande majorité de nos concitoyens désapprouve les personnes éligibles qui font le choix de ne pas se faire vacciner. Au sein même du Parlement, une large majorité s'est dessinée en faveur du passe vaccinal. Je veux saluer, à cet égard, la qualité des débats que nous avons eus en première lecture.

Pendant quatre heures de réunion et de suspension, nous avons cherché à rapprocher nos points de vue de ceux de la majorité présidentielle. Malheureusement, malgré nos efforts et malgré la qualité du dialogue qui s'était instauré, la réaction quelque peu disproportionnée de nos collègues députés députés à un événement extérieur a mis fin à nos espoirs d'aboutir à un consensus, alors qu'un équilibre était en train d'être trouvé sur l'ensemble des dispositions en débat

quelques jours sur la thématique du passe vaccinal. Cela est d'autant plus regrettable que le Sénat, après un débat que l'on peut qualifier de respectueux, d'approfondi

reprendrait à son compte la plupart des points d'accord, certes informels, qui semblaient se dégager lors de la réunion de cette commission. Malheureusement, force est de constater que ce ne fut que partiellement le cas. Il reste, selon nous, deux points saillants de désaccord entre nos deux institutions. En premier lieu, nous réaffirmons notre refus de toute vérification d'identité en cas de doute, dans les cafés, les restaurants, les cinémas, bref, dans les lieux où le passe vaccinal

l'hôtelier ou le restaurateur, car, d'une part, il n'y sera pas contraint et, d'autre part, il s'acquitte déjà d'un devoir assez pénible et chronophage, à savoir la vérification

l'entreprise risquant d'être extrêmement conflictuelle et contentieuse. Nous vous proposerons donc de la supprimer purement et simplement.

deux derniers points à évoquer. L'Assemblée nationale a accepté le système proposé par le Sénat pour les mineurs, qui consiste en un régime unique : il n'y aura pas de passe vaccinal pour les mineurs de 16 ans. de 16 ans. Il est vrai que, en première lecture, le Sénat avait souhaité appliquer cette mesure aux moins de 18 ans, mais nous avions considéré en commission mixte paritaire que cette différence d'appréciation sur l'âge pour l'application

et 18 ans peut décider seul de se faire vacciner sans autorisation parentale, est frappé d'une certaine cohérence. Dernier point et non des moindres : nous n'avons pas pu nous entendre sur la clause d'extinction automatique du passe vaccinal en fonction de critères sanitaires combinés et définis par la loi, clause à laquelle le Sénat était pourtant très attaché. Nous en sommes bien conscients, nous ne pouvons plus introduire dans la loi une date butoir à laquelle le passe vaccinal tomberait de lui-même si le législateur n'était pas de nouveau saisi pour se prononcer sur sa prolongation. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé, à la place, de fixer dans la loi des critères qui, lorsqu'ils seraient réunis, empêcheraient le maintien du passe vaccinal.

Mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera, dans une très large majorité, en faveur de ce texte, sous réserve de la prise en compte des différents points que je viens d'évoquer. Soyez certaine, madame la ministre, que nous travaillons non pas dans un climat d'hostilité, mais dans un esprit de coproduction de la loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat, avec bonne foi et sincérité, pour permettre au passe vaccinal, que nous approuvons, d'être accepté par les Français et d'entrer en vigueur dans les meilleures conditions. La discussion

Ce dispositif qui, si l'on en croit le Gouvernement, devrait encourager les réfractaires à se faire vacciner par lassitude d'être « emmerdés », est devenu, au fil du texte relativement peu lisible. Plusieurs types de passes, en fonction des lieux et du statut vaccinal des personnes, seront mis en place : certains lieux seront accessibles avec le passe sanitaire classique, comme les centres médico-sociaux et les centres hospitaliers, d'autres seront accessibles avec un passe vaccinal, mais des exceptions sont prévues en cas de motif

Plus généralement, l'article 1 instaure une société de contrôle de tous par tous, il restreint les droits des personnes non vaccinées et il donne un sentiment de protection aux personnes vaccinées, lequel peut conduire à l'abandon des gestes barrières dans les endroits confinés soumis au passe. Pour intensifier la vaccination, il faut convaincre et renforcer la politique de l'« aller vers » et non contraindre et multiplier les sanctions. Le taux de vaccination cache d'importantes disparités territoriales. Or ce projet de loi ne traite pas de cette fracture et fait des personnes non vaccinées des citoyens de seconde zone. à d'autres dispositions de cet article, comme le renforcement des modalités de contrôle du passe, le durcissement des sanctions et le prolongement de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion et en Martinique jusqu'au 31 mars Enfin, nos institutions démocratiques sont éprouvées par la multiplication des états d'urgence. Les risques de pérennisation des mesures restrictives prises dans le cadre de ces régimes d'exception sont avérés. Le groupe écologiste s'oppose donc à l'adoption de mesures discriminantes et liberticides et préfère une gestion plus fine pour endiguer l'épidémie : campagne ciblée de vaccination, renfort et soutien financier financier du personnel soignant épuisé, aide et soutien psychologique pour les jeunes, moratoire sur les fermetures de lits d'hôpitaux, généralisation par l'État des capteurs de CO2, mise à disposition des masques les plus efficaces pour les personnes les plus exposées, gratuité des tests ... Votre temps de parole est épuisé, mon cher

un mythe : le passe sanitaire préserverait de la contagion. Il nous aura fallu intervenir à de très nombreuses reprises, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour que le ministre cesse de dire que les lieux soumis au passe sanitaire n'étaient pas des lieux de contagion.

Les sénatrices et les sénateurs sont les représentants des collectivités locales, des territoires. Ils sont en lien direct avec la réalité du terrain, notamment dans le domaine du sport et des infrastructures sportives, lesquelles contribuent

est un amendement de repli.

aucun intérêt pour la gestion de la vague actuelle, autant qu'il en ait un pour les suivantes.

Pour limiter cette atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale, et parce que nos compatriotes n'enfreignent aucune obligation légale de se vacciner, cet amendement vise à rétablir le passe sanitaire tel qu'il résulte de la loi du 31 mai dernier relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans la version qui est actuellement en vigueur. Notre démocratie ne peut fonctionner sous la contrainte déguisée. Les droits fondamentaux, qui garantissent que la liberté est la règle et non pas l'exception,

est à M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à exonérer tous les mineurs, de 12 à 18 ans, du passe vaccinal. Il s'agit de protéger l'ensemble des enfants et des adolescents, qui subissent de plein fouet les conséquences économiques, sanitaires et sociales de la pandémie de covid-19. Le texte prévoit désormais, grâce à l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale, que les mineurs de 12 à 16 ans seront exonérés du passe vaccinal. Nous considérons que cet assouplissement doit également concerner les jeunes âgés de 16 à 18 ans. L'amendement

abandonne donc sa position pour reprendre la mienne ; je ne vais pas pousser la courtoisie jusqu'à abandonner la mienne pour reprendre la sienne. Chiche ! J'ai été tenté de le faire, mais je pense qu'il ne faut pas vider de sa substance le passe vaccinal et faire une loi au rabais- j'ai entendu et lu cette expression. Vous avez raison de faire

des mineurs et considérons qu'à partir de 16 ans, puisqu'on a le droit de se faire vacciner sans autorisation parentale, on doit, comme les adultes, pouvoir utiliser le passe vaccinal en s'en donnant les moyens.

des paramètres objectifs de caducité des dispositifs qui nous sont désormais imposés. Toute l'ironie du rapporteur, que nous pouvons parfois apprécier, n'a pas grande utilité en l'espèce

Les personnes âgées de 12 à 17 ans resteraient quant à elle soumises à l'obligation de présenter un passe sanitaire. La subordination de l'accès aux activités concernées à la présentation d'un passe sanitaire pour les mineurs ne serait possible que dans les départements où les critères prévus pour l'imposition d'un passe vaccinal sont réunis.

certificat de rétablissement. Le problème, c'est que ces derniers sont illisibles en France. Les témoignages sont nombreux, y compris - c'est un comble ! - en provenance de pays membres de l'Union européenne. Les Français de l'étranger ne sont pas les seuls concernés. Alors que la campagne de vaccination bat son plein,

après avoir été infectés alors qu'ils ont besoin de leur passe vaccinal, qu'ils ne peuvent compléter, soit pour rentrer sur le territoire national, soit pour avoir des activités normales une fois sur place. Fonctionnement administratif et règles sanitaires se contredisent, plaçant nombre de nos concitoyens dans une impasse.

La France, en adaptant le passe vaccinal, va s'éloigner du cadre européen du. Ainsi, de nombreux citoyens européens, ou des personnes résidant dans des pays comme le Royaume-Uni ou la Suisse,

Les sanctions prévues apparaissent disproportionnées. L'État, qui se décharge sur des professionnels pour effectuer des missions de contrôle, ne peut leur infliger des sanctions aussi lourdes. Le rôle des exploitants des établissements mentionnés, qui sont déjà fortement touchés par la crise sanitaire, n'est pas de faire respecter les dispositifs du Gouvernement. On ne doit pas les intimider par des mesures répressives. conduit à participer à l'instauration d'une société de contrôle de tous par tous, mais elle transforme substantiellement leur quotidien. Accabler des professionnels déjà acculés par la crise sanitaire et faire preuve de défiance à leur encontre est contre-productif, d'autant que la plupart d'entre eux jouent le jeu avec beaucoup de résilience depuis le début de la pandémie.

de me rendre aux réunions politiques de candidats que je ne soutenais pas, simplement pour me faire une idée de ce que peut être le débat démocratique. Empêcher un citoyen

prévoir dans la loi l'application du passe sanitaire aux réunions politiques, car il estime qu'une obligation générale de cette nature serait susceptible de porter une atteinte excessive au droit des participants de se réunir et d'exprimer leurs idées. L'Assemblée nationale, comme la commission des lois du Sénat, a toutefois souhaité conférer aux organisateurs des réunions politiques la possibilité de décider eux-mêmes de ce qu'ils entendent faire à l'entrée de leurs propres meetings.

est la jurisprudence du Conseil d'État depuis plus d'un siècle. Tout le monde est d'accord avec cette idée. Il est donc logique, dans une période de forte circulation du virus et compte tenu des risques sanitaires, qu'on donne aux organisateurs de manifestations, en clarifiant

Dans ce cas, déposez des amendements de suppression ou de modification significative de l'amendement Larrivé ! Ne laissez pas une telle horreur dans le texte et prenez vos responsabilités ! Le Conseil constitutionnel ne doit pas être la seule institution en mesure de le faire.

Larrivé. Bien évidemment, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller écouter un homme politique. Il serait effectivement malsain que le Gouvernement empêche

je veux parler du rôle saugrenu et extraordinaire donné au conseil de défense et de sécurité nationale. La santé est actuellement considérée comme un domaine réservé du Président de la République, au même titre que la défense, et M. Macron n'est plus seulement le chef des armées : il est aussi le chef de la santé.

Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. » Il semble vraiment très surprenant qu'un tel détournement de la Constitution puisse être banalisé et perdurer. Avec cette pratique, le Parlement, mais aussi le conseil scientifique, et même le conseil des ministres, ont été complètement écartés. Il y a plus grave : tous les comptes rendus de ce conseil de défense sont classés secret défense, c'est-à-dire sont complètement inaccessibles aux citoyens et à bon nombre de parlementaires. nous semble totalement contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont je vous rappelle l'article XV : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

? Mon avis ne peut être que défavorable- je m'en suis longuement expliqué. S'il était adopté, cet amendement créerait un trouble dans la séparation des pouvoirs : c'est au Président de la République de décider ce qu'il entend faire du conseil de défense, qui est mentionné, en effet, dans la Constitution,

Il convient également de rappeler que le droit de vote s'effectue en personne, à l'urne ou par procuration, et d'interdire par conséquent le recours au vote par correspondance ou par le biais de machines électroniques. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement, sur lequel, je n'en doute guère, un compromis saura être trouvé avec les députés.

pour faire obstacle à l'exercice du droit le plus fondamental d'un citoyen français en le soumettant à la production d'un passe vaccinal. Comme vous le savez, mon cher collègue, car vous mettez sans doute un peu de malice dans la présentation réitérée de cet amendement malgré les arguments qui vous ont déjà été opposés, on ne peut demander le passe sanitaire que dans les situations énumérées par la loi. C'est la même chose pour le passe vaccinal : les mêmes règles s'appliquent sans qu'il soit nécessaire de les modifier. ! Par conséquent, vous pourrez revenir sur ce débat autant que vous le voudrez, la règle existe et elle est claire. Toute autre règle serait inconstitutionnelle et les citoyens français, moi le premier, se lèveraient comme un seul homme pour s'y opposer. Permettez-moi

procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

: La parole est à M. Stéphane Ravier. Cet amendement vise à interdire l'obligation du port du masque en extérieur et dans les cours d'école. Ces mesures n'ont aucun fondement scientifique. Ce jeudi 13 janvier, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté préfectoral rendant le masque obligatoire en extérieur à Paris. Le tribunal administratif de Versailles a rendu une décision similaire la veille, mercredi 12 janvier, arguant d'« une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée [ ...] à la liberté individuelle ».

recevant du public et dans les écoles. Le Sénat avait adopté cet article, contre l'avis de la commission, pour rappeler au Gouvernement ses obligations à l'égard des collectivités locales. La commission estime

Nous apprenions, le 7 janvier 2022, que le Gouvernement avait retiré la demande d'autorisation formulée auprès de la CNIL pour l'entrepôt de données de santé dit Health Data Hub. Avec

publique prévoit que, « lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé », y compris psychiatrique, donc, « il est proposé au patient de désigner une personne de confiance

privés d'une loi sur la santé mentale pourtant promise par plusieurs gouvernements, le refus de tout amendement sur cet article qui fait figure d'intrus dans ce projet de loi renforce la désagréable impression d'un débat interdit. On me dit que cet amendement est secondaire par rapport aux autres articles Oui, cet article n'a rien à faire là ; mais non, l'encadrement de la contention et de l'isolement en psychiatrie n'est pas un sujet secondaire. Je vous demande, mes chers collègues, de le réaffirmer

ce qui est une grave erreur. Il nous revient, à nous, législateurs, de ne pas sacrifier la loi sur l'autel misérable de la politique politicienne. Revenons au projet de loi. Cette obligation vaccinale qui ne dit pas son nom pourrait avoir des effets négatifs à long terme. La lecture

Une nouvelle fois, l'exécutif cède à la panique et empiète toujours davantage sur nos libertés, marginalisant ainsi toute une partie de la population.

Je reste persuadée de l'importance et de l'efficacité du vaccin, mais son utilisation doit être proportionnée et rationalisée, comme le rappelle la Défenseure des droits dans son dernier avis. Je voterai donc contre ce texte. La

à une position claire. Pour nous, seules les forces de l'ordre peuvent

mon sentiment, c'est que nous venons d'assister à une folie. En tant que parlementaire, en tant que médecin, j'ai en tête de Stefan Zweig : « Je [ne suis] plus qu'un médecin, un homme de dévouement, d'intuition et de science. »

et prendre son temps, comme si nous pouvions encore passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines à discuter. C'est pourtant ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.